Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Monsieur le ministre, j'avais prévu depuis plusieurs jours de vous interroger sur les tensions grandissantes dans les relations entre la police et les citoyens. J'avais d'ailleurs

Cela étant, je veux aussi, bien sûr, affirmer avec force qu'il n'est pas possible de laisser toute une institution républicaine- la police nationale et ses agents -salie par les comportements intolérables d'une infime minorité. Nous savons l'importance des missions exercées par nos forces de l'ordre. La sécurité est en effet le premier des droits, notamment pour nos concitoyens les plus fragiles. C'est également la garantie de notre liberté.

manque de reconnaissance, pression liée au contexte politique mouvementé ou au terrorisme. Dans ce cadre explosif, la dégradation des relations entre la police républicaine et nos concitoyens, qui n'a cessé de s'aggraver durant les semaines de confinement, a été malheureusement trop souvent reléguée au second plan. C'est pour cette raison, mais aussi du fait du contexte international, que la manifestation d'hier devant le tribunal de Paris a trouvé un écho important. Je condamne bien entendu fermement les violences qui sont survenues à la fin de ce rassemblement. Il est pourtant impératif, voire urgent,

pour permettre aux forces de l'ordre de travailler sereinement ? Pouvez-vous nous préciser si le stock de plusieurs millions d'heures supplémentaires dues aux agents va enfin être payé ?

Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, d'une décision et d'une sanction.

attentifs, en nous engageant, pour répondre à votre question, auprès de la police et de la gendarmerie. Depuis 2017, le budget de la police et de la gendarmerie a augmenté de 1 milliard d'euros, ce qui est significatif. Depuis 2017, nous avons lancé un programme de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires pour tous les services, qu'il s'agisse du renseignement, mais aussi de la police de sécurité du quotidien. Monsieur le sénateur, pour clore mon propos, je vous renvoie non pas aux commentaires, mais à la réalité d'analyses sérieuses. Récemment, l'université Savoie Mont-Blanc a travaillé sur le rapport entre les citoyens et la police : 48 134 personnes ont été interrogées dans ce cadre, et 85,3 % d'entre elles ont une opinion très positive ou positive de la police nationale et de la gendarmerie. C'est cela la réalité, ce ne sont pas les commentaires médiatiques. La réalité, elle ne se fait pas sur les réseaux sociaux

Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Le groupe automobile Renault vient d'annoncer la suppression de 4 600 emplois dans notre pays. Bien au-delà des effets de la pandémie en cours, nous payons là le choix des délocalisations massives vers les pays à bas coûts pratiquées ces deux dernières décennies. Les menaces pesant sur l'avenir de certains sites suscitent, on l'a constaté, d'énormes inquiétudes dans les territoires concernés : Maubeuge, malgré les annonces récentes, mais sans réelle garantie au-delà de 2023, Choisy-le-Roi, Flins, Caudan ou encore Dieppe. Le chiffre d'affaires de Renault fut de 55 milliards d'euros en 2019. L'État actionnaire a annoncé l'octroi d'une garantie publique de 5 milliards d'euros. M. Jean-Dominique Senard, président de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, a déclaré sur France Info, lundi soir, que cette garantie ne s'accompagnait pas de « contraintes difficiles ». Madame la secrétaire d'État, quelles contraintes allez-vous imposer au groupe Renault ?

faire prendre des engagements à Renault. Je vous rappelle que le prêt garanti par l'État n'était pas encore signé hier. Ce sont ces engagements-là que nous prenons en donnant cette garantie. Jean-Dominique Senard a été très clair. Premièrement, Renault est en grande difficulté, je crois que

de réduction des coûts. Ce plan concerne certes la France, mais aussi d'autres pays. La question est non pas de délocaliser des productions, mais de faire face à une diminution du nombre d'achats de voitures. Renault peut produire 5 millions de voitures ; malheureusement, elle n'en vendra peut-être que 3 millions, 3,2 millions ou 3,4 millions cette année. On voit bien là l'écart de production par rapport aux capacités industrielles.

à ce site et à continuer d'y maintenir des activités. Dernier point, Renault s'est engagé à relocaliser des productions en France, notamment en ce qui concerne la traction électrique, et à investir dans la batterie électrique, ce projet européen qui est si important pour notre industrie automobile. La parole Madame la secrétaire d'État, les sites de production des modèles Twingo, Clio et Dacia sont implantés en Turquie, en Roumanie et en Slovénie. Ces usines tournent sept jours sur sept et sont surchargées. Il faut décider de relocaliser la production de 300 000 de ces véhicules, afin d'apporter de la commande aux sites de production de notre pays. dans le même temps de réorienter la production vers des modèles hybrides, électriques et thermiques à prix modique, afin d'accélérer la transition énergétique. Cela pose aussi en creux la question du pouvoir d'achat. Personne ne comprendrait que l'argent public ne serve qu'à accompagner les suppressions d'emplois. Notre industrie automobile mérite un autre développement, un autre avenir et un engagement fort et déterminé de l'État actionnaire !

C'est dans un contexte de chute brutale des rentrées fiscales que le Premier ministre a annoncé ce vendredi une garantie des recettes pour les outre-mer : 110 millions d'euros pour les communes ; 40 millions d'euros pour les régions et collectivités uniques. Ce sont des mesures que nous avions très tôt proposées et que nous sommes aujourd'hui satisfaits de voir actées. Toutefois, vous nous proposez une enveloppe de 150 alors que notre collègue sénateur Georges Patient, auteur d'un rapport sur le sujet, parle pour sa part de 200 millions d'euros, d'autres experts avançant même la somme de 240 millions d'euros. Nous sommes donc encore manifestement très loin du compte ! Outre ces premières mesures, des experts, mandatés par Bercy, ont également commis un rapport qui vous propose de remplacer l'octroi de mer par des points de TVA supplémentaires. Madame la ministre, évitons-nous ce débat déstabilisant et anxiogène. Nos collègues vous demandent d'écarter cette option mortifère, qui n'a fait l'objet d'aucune consultation. Au lieu de réformer l'octroi de mer, ils vous proposent de rattraper le niveau des dotations de péréquations : versez, dès cette année, les 85 millions d'euros qui font défaut aux outre-mer.

la crise sociale à laquelle feront face les départements et de supprimer les contrats du pacte de Cahors. Madame la ministre, quelle réponse pouvez-vous faire à ces légitimes demandes ?

l'effort est à la hauteur des besoins. Vous avez évoqué un certain nombre d'évaluations : ce ne sont que des évaluations. Nous nous sommes effectivement mis d'accord avec l'ensemble des collectivités pour les réaliser, mais nous avons aussi décidé que le rendez-vous serait fixé à la fin de l'année.

Bien sûr, il faut une évaluation ; celle-ci a été chiffrée : le rapport du député Cazeneuve nous a servi de base, mais les débats continuent, et nous aurons l'occasion d'en reparler.

d'une forme d'octroi de mer ou de taxes sur les carburants. Par conséquent, c'est la première fois que l'on embrasse la totalité des territoires ultramarins et que l'on est aux côtés de tous les territoires.

Je tiens tout de même à souligner que l'urgence est de prévenir tous les risques d'incapacité budgétaire, en permettant aux collectivités d'outre-mer de sortir de l'ornière et de retrouver des marges de manoeuvre. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que l'investissement et l'économie des outre-mer dépendent essentiellement de la commande publique. Nous comptons sur vous pour aller

ministre de l'intérieur. C'est un parlementaire quelque peu décontenancé qui vous interroge, monsieur le ministre, à propos de la reconnaissance des élus locaux sans étiquette.

En 2010, le Conseil d'État avait rejeté le recours formulé contre l'impossibilité pour les élus d'être reconnus et classés « sans étiquette ». Ce combat ancien, nous pensions le partager avec vous, monsieur le ministre. Lorsque mon collègue Dany Wattebled vous a interrogé sur votre volonté d'intégrer cette rubrique dans les documents des élections municipales de 2020, vous sembliez ouvert à la discussion- « à notre écoute », pour reprendre l'expression que vous aviez utilisée ! Votre circulaire tant décriée du 10 décembre 2019 apportait un début de réponse, en supprimant le nuancement politique pour les candidats dans les communes de moins de 9 000 habitants. La circulaire a été suspendue par le Conseil d'État. Celle du 3 février a rabaissé le seuil aux communes de moins de 3 500 habitants, hors chefs-lieux de canton. Nous n'avons pas crié victoire, mais nous pensions que le concept d'élu « sans étiquette » était acquis. Or, depuis quelques jours, j'ai un horrible doute. Certains maires m'ont fait part de leurs déceptions et de leurs interrogations en remplissant le document de déclaration des résultats. Dans celui-ci, leur étiquette politique leur est demandée, y compris dans les communes de moins de 3 500 habitants. Ma question est donc claire votre circulaire du 3 février 2020 s'adresse-t-elle aux déclarations de candidature et aux documents de résultats des élections ou s'adresse-t-elle uniquement aux seules déclarations de candidature ?

de la représentation nationale ou dans les partis politiques, mais qui correspond à l'expression des maires ne voulant pas se reconnaître dans telle ou telle étiquette politique. L'instruction que je donne au moment où je vous réponds et que je confirmerai si c'est nécessaire est la suivante : les préfets doivent être à l'écoute des maires désignés par le conseil municipal ; la qualification « divers » relève de leur appréciation, et nous devons

Il se développe une réelle impunité, la violence et la menace ayant depuis longtemps pris la place de la loi et de forces de l'ordre de plus en plus spectatrices de situations qui leur échappent. L'autorité de l'État, à leurs yeux, n'est plus qu'un mot. À force de laisser faire, d'excuser et de ne rien faire, l'État a perdu le contrôle. Nous récoltons les fruits amers de nos renoncements. L'une de nos collègues, Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice du Val-d'Oise, est aujourd'hui victime de cette violence et de ces intimidations, qui touchent tous ceux qui représentent l'État ou les pouvoirs publics. n'acceptent pas une décision prise par la mairie de sa ville ont choisi de s'en prendre à notre collègue. Vendredi dernier, elle a été copieusement insultée. Lundi, un groupe d'une quarantaine de personnes a fait le siège de son domicile, l'empêchant de sortir de chez elle, allant jusqu'à la menacer de s'en prendre à sa mère âgée, qui habite un quartier d'HLM de la ville. Avant que ce groupe, qui déambulait dans la ville, n'arrive devant son domicile, la police municipale avait pourtant prévenu la police nationale de ses intentions. Hier, ce même groupe a recommencé sa bruyante déambulation, bloquant la circulation, s'installant sur plusieurs giratoires, pour finir par revenir devant le domicile de notre collègue et y proférer des menaces. Aujourd'hui notre collègue ne peut plus circuler librement dans sa ville. Hier, une manifestation interdite en plein état d'urgence sanitaire, qui a réuni 20 000 personnes devant le palais de justice de Paris, a dégénéré. La justice y était accusée de couvrir la gendarmerie dans un dossier que, hélas, je ne connais trop que Quelle inversion des valeurs ! Ce sont désormais les voyous qui tiennent la dragée haute aux représentants de l'État, aux forces de l'ordre. L'impunité leur donne toute leur force. Ces voyous savent qu'ils ne risquent rien : la politique de votre gouvernement est de vider les prisons. Monsieur le ministre, où est l'État ? Qu'est devenue l'autorité de l'État ?

pour garantir sa liberté d'expression, sa liberté de dire et de combattre, comme elle le souhaite, comme elle le veut, non pas seulement parce qu'elle est sénatrice- ce serait déjà une excellente raison -, mais tout simplement parce que, dans ce pays, nous devons garantir la liberté d'expression de chacun. Néanmoins, je ne peux pas vous laisser dire que les voyous voyous tiennent aujourd'hui la dragée haute à notre police où à notre gendarmerie. Chaque jour, chaque nuit, chaque fois que la police est appelée, elle vient. Chaque fois, elle intervient. On a beaucoup évoqué ces derniers jours, comme hélas depuis de longues années, la question des violences urbaines. Comme vous, je les dénonce, mais je fais en sorte que la police soit renforcée. J'évoquais notre décision de procéder à 10 000 recrutements, qui sont nécessaires pour que nous soyons présents partout, y compris dans les quartiers. Et nous sommes présents partout, y compris dans les quartiers N'analysons pas les événements médiatiques comme une ligne ou une tendance en matière de violence urbaine. Par rapport à l'année dernière, nous nous situons sur une constante, y compris d'ailleurs pendant la période du confinement, excepté en Île-de-France, où nous avons connu une augmentation significative des incidents- cela n'a pas été le cas sur l'ensemble du territoire national.

c'est un combat que nous devons mener, pas seulement, monsieur le sénateur, par l'interpellation, mais aussi par la prévention et par la présence policière. Je ne souhaite pas opposer la nécessité d'une police de sécurité du quotidien, qui s'appuie sur le travail des élus pour porter une ambition pour les quartiers les plus difficiles de notre pays,

il a rappelé les garanties sociales associées audit prêt, telles que le maintien de l'emploi et de l'activité industrielle sur le site de Maubeuge au-delà de 2023. Ces garanties sont rassurantes,

ce prêt intervient quatre jours à peine après l'annonce d'un plan de restructuration et la suppression de 4 600 emplois en France, pour un fleuron industriel national. Ce prêt intervient également sept jours après la présentation d'un plan de soutien massif à l'industrie automobile, qui devait être la rampe de lancement d'une souveraineté économique retrouvée ... Ce plan, et plus globalement la stratégie de l'État actionnaire, parviendront-ils, au pire, à empêcher la désindustrialisation hexagonale, au mieux, à permettre la relocalisation dans notre pays d'une partie de la production ? Et si oui, laquelle ? Enfin, entre un plan de soutien à l'automobile, qui se veut un véritable pacte, et ce nouveau prêt,

vous-même, monsieur le ministre, avez présenté la carte de la seconde phase du déconfinement. Si presque toute la France est passée au vert, Mayotte et la Guyane sont, avec l'Île-de-France, désormais classées au niveau de vigilance orange. Mayotte est le territoire d'outre-mer le plus touché par le Covid-19. Plus de 1 993 cas y ont été identifiés et 24 décès sont à déplorer. En Guyane, le virus s'est considérablement propagé ces dernières semaines, pour atteindre 517 cas positifs, dont 1 décès. cette progression de l'épidémie n'est pas sans lien avec l'inquiétante situation sanitaire de son voisin brésilien. L'État d'Amapá, à lui seul, compte en effet près de 9 900 cas positifs, 222 décès et un système de santé totalement saturé. Le virus ne s'embarrassant pas des frontières, les communes de Saint-Georges de l'Oyapock et de Camopi sont rapidement devenues les deux premiers clusters de Guyane. En réponse, la mobilisation récente de la réserve sanitaire est venue renforcer une campagne massive de tests déployée dans l'Est guyanais, campagne qui reste cependant limitée au sol français. À Mayotte, ces actions rapidement mises en place commencent à porter leurs fruits, et, hormis le cluster important récemment découvert à la prison de Majicavo, la situation semble se stabiliser. Mais en Guyane, considérant la porosité de la frontière, nous pouvons nous interroger sur l'efficience de mesures qui se limiteraient à la seule rive française de l'Oyapock. Il y va de la protection de la population de l'Est guyanais, bien entendu, mais pas seulement, puisque la circulation du virus s'intensifie dans l'ensemble du territoire. Pouvez-vous nous dire comment le Gouvernement entend faire évoluer la stratégie sanitaire en Guyane, au regard de la poussée de l'épidémie au Brésil ? Un dispositif de coordination et de mutualisation des moyens ne pourrait-il pas être mis en oeuvre, dans le cadre de la coopération transfrontalière ? La

Il devrait, dans ces conditions, se faire un devoir de laisser de côté toute attitude qui conduirait à privilégier les représentants d'une chambre plutôt que ceux d'une autre, ou, pire, à favoriser sa famille politique. Alors Alors que les déplacements se multiplient, les modalités de leur organisation nous laissent désormais songeurs. Ainsi les préfets précisent-ils par écrit que, dorénavant, compte tenu des conditions sanitaires et du maintien des gestes barrières, le choix a été fait qu'un seul député représenterait l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs,

de la représentation nationale n'est pas propre à mon département. Mes collègues de Saône-et-Loire, des Yvelines, de la Haute-Garonne, de l'Oise et d'autres départements ont vécu ces derniers jours exactement la même situation.

S'agit-il alors d'une instruction gouvernementale qui viserait à écarter les sénateurs ? Aucun parti ne peut être la République à lui seul

Cela se comprenait aisément, compte tenu de la situation particulière que nous vivions. Depuis le 11 mai, cette situation particulière perdure malgré tout, même si les conditions sanitaires se sont améliorées au fur et à mesure du temps. Au fond, depuis le 11 mai, ce qui doit dominer,

Je m'exprime au nom du groupe socialiste, plus particulièrement au nom de mes collègues de Seine-Maritime et du Val-de-Marne. L'État a garanti un prêt de 5 milliards d'euros à Renault, tandis que ce groupe annonçait un plan d'économie prévoyant 4 600 suppressions de postes en France et la restructuration de 6 usines. Nous nous félicitons que la colère des salariés de Maubeuge

d'autant plus que d'autres sites sont en sursis. À Dieppe, il n'y a aucune garantie de la pérennité de l'usine Renault Alpine. À Choisy-le-Roi, la fermeture de ce modèle d'économie circulaire est une aberration.

le permettre. Il faut en effet rompre avec trente ans de délocalisations ! Nous avons besoin d'un État qui favorise un large investissement et insuffle une stratégie pour la filière automobile et la réindustrialisation du pays, qui accélère la recherche-développement afin de favoriser l'innovation au service de l'écologie. L'industrie, particulièrement le secteur automobile, doit se verdir pour respecter l'accord de Paris et l'engagement de mettre fin à la vente de véhicules thermiques. Madame la secrétaire d'État, l'État, actionnaire majoritaire de Renault, va-t-il imposer des exigences écologiques ? Les aides publiques aux entreprises seront-elles enfin conditionnées au respect de critères sociaux et environnementaux ?

Dans ce contexte est paru, le 23 avril dernier, un décret visant à réquisitionner cinq produits d'anesthésie en pénurie. Depuis lors, la situation sur le terrain est illisible. Les pharmacies hospitalières ne peuvent plus commander ces produits, puisque l'État en détient désormais le monopole d'achat et de livraison, la gestion en local se faisant les ARS. Le but était de rendre prioritaires les établissements les plus touchés par l'épidémie. Les faibles taux d'approvisionnement imposés ont créé de très fortes tensions dans les territoires. Ces dernières semaines, nombreux ont été les établissements de soins insuffisamment approvisionnés. Beaucoup d'interventions ont dû être décalées. Certains hôpitaux sont rationnés, d'autres sont livrés, mais sans que l'on sache comment est faite Des alternatives dégradées de prise en charge sont mises en place ; c'est un réel recul, avec des risques pour les patients. Une nouvelle crise sanitaire se profile. La situation est urgente dans certains départements. Les pharmaciens hospitaliers, en lien direct avec les besoins, sont dans un carcan, ne permet ni la réactivité ni la souplesse qui sont nécessaires, pour ne pas dire vitales. Faute de transparence et de dialogue sur la gestion, les disparités se creusent, l'équité face aux soins est mise à mal. Même la perspective d'une éventuelle seconde vague ne saurait justifier cette situation. Monsieur le ministre, le stock national est-il reconstitué, comme cela semblerait logique ? Quelles sont les clés de répartition actuelles qui créent des disparités délétères ? Les besoins sur le terrain pour les patients autres que ceux atteints du Covid sont réels. Quand pensez-vous mettre un terme au contingentement actuel et redonner la main aux acteurs de terrain dans les établissements de santé ?

Le problème n'est pas nouveau, puisque la fabrication des molécules de médicaments est aujourd'hui délocalisée à 80 %. Les stocks de nombreux traitements dépendent de réseaux de distribution internationaux, et certains médicaments, notamment des génériques, sont fabriqués uniquement en Inde ou en Chine.

et complexe. Toutefois, il serait possible d'envisager un rapatriement progressif sur le territoire français et européen. La fabrication de molécules majeures, par exemple celles qui sont utilisées dans le traitement du cancer ou de longues maladies, doit faire partie des priorités, tout comme la production de médicaments génériques, aujourd'hui sous-traitée à 100 % et qui devrait, au moins en partie, être relocalisée sur le sol français. N'oublions pas que cette pénurie a créé de graves tensions lors de la prise en charge des maladies liées au Covid. En mars dernier, les hôpitaux européens, notamment ceux de Paris, ont alerté les pouvoirs publics sur le manque de médicaments essentiels dans les unités de soins intensifs et de réanimation. Ce type d'alerte doit impérativement être pris au sérieux si l'on veut éviter de reproduire les mêmes erreurs.

En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de la loi du 23 juillet 2010, adoptées pour son application, la commission des finances a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable, par 9 voix pour, aucune voix contre et 4 bulletins blancs, sur la nomination de Mme Isabelle Falque-Pierrotin aux fonctions de président du collège de l'Autorité nationale des jeux. avons terminé avec le débat sur le thème : « Quelles nouvelles politiques publiques à destination de la jeunesse afin d'aider ces publics particulièrement exposés dans la prise en charge des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire ? » Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes,

Je partirai d'un postulat, sans lequel il me semble impossible de débattre et de construire de nouvelles politiques pour la jeunesse ; il s'agit d'affirmer et, surtout, d'inscrire dans les faits que, comme Jean Jaurès le disait au sujet de la nature humaine, nous devons faire un large crédit à notre jeunesse. Faire confiance à la jeunesse et la soutenir, cela relève de l'urgence, car, si les jeunes sont heureusement les moins touchés par la pandémie, ils sont malheureusement en première ligne de la crise économique et sociale dont nous redoutons l'ampleur. Si nous avons voulu ce débat sur le thème : « Quelles nouvelles politiques publiques à destination de la jeunesse ? », c'est que nous estimons que la situation sociale n'a pas été suffisamment prise en compte par le Gouvernement, alors qu'il faut anticiper et aider les plus fragiles à traverser la crise. L'augmentation du chômage nécessite des mesures fortes pour empêcher de nombreux jeunes de basculer dans la précarité. La crise sanitaire que nous traversons se double en effet d'une crise économique et sociale, dont nous ne pouvons que redouter les effets dévastateurs. Il faut faire, là aussi, jouer la solidarité nationale.

Nous estimons que l'État, garant de la solidarité nationale et de la justice sociale, doit intervenir et mettre en oeuvre des politiques publiques ancrées dans le quotidien des jeunes. Quel sens, quelle valeur donner à ces politiques publiques qui se définissent avant tout comme la réduction des écarts, c'est-à-dire l'attention aux plus fragiles, aux plus déshérités pour lutter contre les inégalités sociales et spatiales ? Quelle place accorde-t-on, dans notre politique d'emploi et de logement et dans notre système de protection sociale, à notre jeunesse, qui est particulièrement exposée aux conséquences de la crise sanitaire ? En effet, les jeunes de 18 à 25 ans, qui constituent 30 % des salariés des entreprises durement touchées par le confinement- restaurants, commerces et centres de loisirs -, ont été privés de revenus, alors que 670 000 étudiants en dépendent pour leurs besoins les plus essentiels- alimentation, logement, habillement -et que 20 % des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. 30 % des 18-22 ans pensent ne pas trouver de cet été et 15 % d'entre eux ont vu leur stage être annulé, sans solution de rechange. Nombreux seront ceux qui ne pourront pas financer leurs études ou payer leur loyer ... Comment donner confiance à cette jeunesse, alors que le logement leur devient inaccessible et que le Gouvernement annonce une récession de 11 % ? Mes collègues Corinne Féret, Claudine Lepage et Viviane Artigalas reviendront sur plusieurs points, notamment sur la question de l'autonomie financière des jeunes-

surtout renoncer à la réforme, prévue en 2020 et déjà reportée quatre fois, de l'APL, qui fera perdre l'allocation à 600 000 personnes, dont près de 300 000 jeunes. Est-il raisonnable de continuer dans cette voie, alors que les jeunes sont particulièrement visés par ce dispositif ? Ce sera insupportable. Annulez cette réforme vous l'avez déjà reportée quatre fois, encore un petit effort ... Si cette précarisation frappe durement les jeunes en général, elle frappe encore plus durement les jeunes de nos quartiers.

Si la crise de 2008, qui a affecté la finance et les services, a eu un impact sur la jeunesse, l'effet est, cette fois, plus concentré sur les moins qualifiés, sur les bas salaires et sur les plus jeunes, autant de facteurs qui conditionnent la bascule dans la pauvreté, comme en ont témoigné les files d'attente de la faim. Face à l'urgence de la situation, il nous faut répondre, tout de suite, avant le mois de septembre. C'est un discours positif et volontaire qu'il faut tenir à la jeunesse. La richesse de la jeunesse, nous devons la reconnaître et la valoriser ; d'ailleurs, nombre de jeunes ont travaillé pour les autres pendant cette crise. Au regard de la réalité sociale et économique, le pourcentage de jeunes en insertion devrait être quatre, voire cinq fois plus élevé. Mme Muriel Pénicaud nous l'indiquait la semaine dernière, seuls 16 des jeunes des quartiers ont des emplois aidés. C'est ainsi que nous donnerons corps au principe d'équité, sans lequel nulle justice ne peut être vécue ni même perçue. J'ai déjà évoqué la réactivation des contrats aidés, qui peut constituer un levier de soutien fort et rapidement mobilisable : des jeunes apportant leur savoir et leurs compétences à nos communes et à nos associations, et trouvant, par ce biais, une première insertion dans l'emploi, encadrés par des adultes.

en avait plus que 130 000. Oui, leur remise en cause drastique et brutale a signifié non seulement le retour à la précarité pour nombre de jeunes, mais encore la fragilisation du monde associatif.

Monsieur le secrétaire d'État, au regard des besoins existants dans les écoles et les collèges des quartiers, et considérant la nécessité de donner un avenir aux jeunes de ces quartiers, le Gouvernement compte-t-il réactiver les contrats aidés et revenir sur le jugement péremptoire consistant à estimer qu'ils sont trop coûteux et peu utiles ?

Cela aiderait la jeunesse, mais aussi nos enfants et les associations. Il s'agit là d'un véritable défi éducatif et démocratique. Il y a une urgence, une urgence économique et sociale pour les jeunes ; de la jeunesse dépend notre avenir collectif.

engagée, et je veux, comme vous, rendre hommage à leur dynamisme, à leur civisme et à leur sens indéniable de l'engagement collectif. Loin des idées reçues, nous pouvons être fiers de cette génération qui, pendant la crise sanitaire, a su mobiliser une formidable Parmi les 300 000 personnes qui se sont spontanément portées volontaires au travers de la plateforme de la réserve civique, 40 % avaient moins de 30 ans ; 58 000 jeunes en service civique ont transformé leur mission pour contribuer à l'effort national contre la pandémie, et l'on ne compte pas les jeunes qui se sont engagés bénévolement, dans leur quartier, au pied de leur immeuble, pour subvenir aux besoins

venir. Pendant la crise sanitaire, le Gouvernement a répondu, vous le savez, avec une force sans précédent aux drames économiques et sociaux. Notre action pour tous les Français a directement bénéficié aux jeunes ; quand on prend des mesures de soutien à l'activité économique, à l'emploi et aux entreprises, on prend indirectement des mesures de soutien aux jeunes, et l'ensemble des dispositifs que nous avons pris permet de limiter les dégâts sur le monde économique et donc sur l'emploi veux également mentionner les règles régissant le chômage et l'activité partiels, règles qui ont été assouplies pour protéger les demandeurs d'emploi en fin de droits, les intérimaires et les travailleurs saisonniers en faisant perdurer leurs droits au-delà du confinement. Je pense aussi aux jeunes parents, obligés de garder leurs enfants, qui ont bénéficié d'un système exceptionnel d'indemnités Je veux également citer les mesures de solidarité avec les personnes précaires et l'aide de 150 euros qui a été versée à 4 millions de familles pauvres ou modestes, à laquelle s'est ajouté un montant de 100 euros supplémentaires par enfant. Cela représente un effort global de 900 millions d'euros, largement fléché vers les enfants et vers les jeunes. Nous avons également agi directement et spécifiquement en direction de la jeunesse. La principale mesure a consisté en une mobilisation de 150 millions d'euros, sous la forme d'une aide exceptionnelle de 200 euros pour 800 000 jeunes, destinée à compenser la perte de revenu liée à l'arrêt temporaire d'un stage, d'un apprentissage ou d'un étudiant. Cette prime sera versée

et scolaires (Crous) ont pris la décision de n'exiger aucun préavis des étudiants qui ont décidé de mettre fin à leur bail en résidence étudiante, afin de leur éviter un surcoût inutile. Nous avons prolongé les dispositifs de l'aide sociale à l'enfance (ASE) pour les enfants atteignant

d'euros. Il faut maintenant penser à l'après-crise, vous l'avez dit. À ce titre, quatre grands axes de travail, sur lesquels je reviendrai à l'occasion des questions, nous mobilisent. Tout d'abord, il faut lutter contre le décrochage scolaire, notamment dans la voie professionnelle, parce qu'aucun jeune ne doit être désoeuvré ni se sentir laissé pour compte. Ensuite, nous devons maintenir la dynamique engagée par notre gouvernement sur la formation et sur l'apprentissage ; forts de de nos réussites, et parce que le contexte nous y incite, nous devons aller plus vite et plus fort. En outre, il est nécessaire de faciliter l'accès à l'embauche ; le marché du travail risque de se durcir, nous devons aider les entreprises à embaucher des jeunes et aider les jeunes à accéder à l'emploi. Enfin, il convient d'agir pour lutter contre la précarité des jeunes face

Nous avons mobilisé 15 milliards d'euros pour la formation de 1 million de jeunes et de personnes peu qualifiées. Nous avons développé des solutions multiples de la deuxième chance et de lutte contre le décrochage scolaire, notamment pour les jeunes

Je réfléchis en ce moment à des dispositifs de soutien à l'emploi associatif, en lien avec le volet associatif de mes responsabilités, mais cela pourrait tout à fait se croiser avec la préoccupation de l'emploi des jeunes. Il y a là des ponts intéressants à construire dans les semaines à venir ; en tout cas, j'y suis tout à fait disposé. Je suis sûr que surgiront de nos débats des idées fructueuses pour les mois à venir. je vous remercie Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

constituent une population fragile, combien ils sont vulnérables face au fléau du chômage, combien ils sont, plus que d'autres, susceptibles de tomber dans le découragement et la crainte de ne pas parvenir à s'insérer dans le monde du travail. Parmi les dispositifs destinés aux jeunes, le service civique semble particulièrement pertinent pour favoriser l'intégration, pour créer le lien social et pour faire acquérir à nos jeunes des compétences, qu'ils peuvent par la suite valoriser dans le cadre d'une première embauche. Cette année, le service civique a 10 ans et son petit frère, le service national universel, fête, lui, sa première année d'expérimentation. Ma question est la suivante : peut-on dresser un bilan du service civique depuis son instauration et, surtout, que peut-on dire du service civique et de son rôle au cours de cette période de confinement ? Peut-on envisager un élargissement de ce dispositif, ce qui impliquerait, vous l'aurez compris, monsieur le secrétaire d'État, d'augmenter son budget ? Autrement dit, le service civique peut-il être un élément structurant de l'indispensable accompagnement des jeunes dans l'ère post-Covid-19 ? Enfin, j'aimerais attirer votre attention, monsieur le secrétaire d'État, sur les jeunes en situation de handicap, qui représentent à peine 3 % des volontaires du service civique. Au regard de la précarité et de la fragilité accrue de ces jeunes, un renforcement de leur accès au service civique

qui fête, vous l'avez dit, ses 10 ans cette année. Nous avions prévu un grand moment réunissant 1 000 jeunes du service civique, qui devait se tenir à la fin du mois de mars. Évidemment, nous avons dû le reporter, mais le service civique est un magnifique dispositif, et il faut le dire.

conçu comme une brique supplémentaire de l'insertion dans l'emploi, mais il s'est imposé comme un moment permettant aux jeunes de prendre confiance en eux, de découvrir des choses, de développer un certain nombre de compétences, notamment des savoir-être, et d'être valorisés ensuite dans une logique d'insertion dans l'emploi. En effet, beaucoup d'entreprises et de représentants du patronat estiment aujourd'hui que le service civique est devenu une forme de label sur un CV ; ils considèrent qu'un jeune

jeunes feront une mission de service civique. Il faut continuer de le faire croître et, pour répondre à votre question, cela peut constituer l'une des réponses à la crise que nous vivons,

j'accorde une grande importance à la qualité des missions : je l'ai souligné dès ma prise de fonctions, il ne faut pas tomber dans la substitution à l'emploi ni dans des missions qui ne serviraient qu'à occuper les jeunes. Si le service civique a fonctionné, c'est parce que les jeunes sont utiles et se sentent tels. Il faut évidemment poursuivre dans cette voie, et c'est ce à quoi nous travaillons.

permet d'aller plus loin en matière d'insertion. Il est étonnant de voir le nombre d'associations qui se chargent d'accompagner le handicap

On annonce, malgré des aides de l'État, 4 600 suppressions d'emploi. Vous imaginez bien que ce sont autant de débouchés en moins pour nos jeunes dans des régions industrielles comme les nôtres, où la situation est déjà très difficile

Monsieur le secrétaire d'État, alors que 750 000 jeunes s'apprêtent à finir leurs études, leur insertion sur le marché du travail s'annonce particulièrement difficile cette année. l'emploi des cadres (APEC) observe une chute de 69 % des offres d'emploi destinées aux jeunes diplômés par rapport à l'année dernière. Le plan global en faveur de la jeunesse annoncé par le Gouvernement est, à cet égard, très attendu.

De nombreux centres de formation sont menacés de fermeture par la crise. En effet, depuis la dernière réforme, le financement de ces centres dépend du nombre de contrats signés. Or peu de PME et de TPE sont prêtes à signer de nouveaux contrats à la rentrée, compte tenu des incertitudes économiques qui pèsent sur de nombreux secteurs, en particulier celui de l'hôtellerie et de la restauration, qui emploie, chaque année, de nombreux apprentis. Monsieur le secrétaire d'État, dans le contexte actuel, ne serait-il pas souhaitable, d'une part, de revoir transitoirement les règles de financement des centres de formation, en calant les sommes attribuées par les opérateurs de compétences sur les effectifs de 2019, de faciliter les entrées et sorties des élèves apprentis dans le dispositif d'apprentissage, afin de laisser davantage de temps aux entreprises de se remettre à flot sans pénaliser les jeunes, qui sont de plus en plus nombreux à souhaiter se former par cette voie

posez la question de l'apprentissage, qui, comme je l'ai dit dans mon intervention liminaire, est une très grande priorité pour le Gouvernement. Grâce à la mobilisation absolue de Muriel Pénicaud, nous avons enfin réussi à faire, pour notre pays, ce que beaucoup ont cherché à faire depuis

faut donc que, pour cette année 2020, nous soyons en mesure d'accueillir au moins autant de jeunes en apprentissage que l'an dernier. Je pense que c'est un objectif raisonnable que nous pouvons nous fixer. aura lieu une réunion très importante entre les partenaires sociaux et le Président de la République, pour aborder un certain nombre d'enjeux qui ont trait au marché du travail et à l'emploi. La question de l'apprentissage sera centrale dans ces discussions. Il m'est compliqué de faire des annonces : celles-ci interviendront, par définition, après l'échange avec les partenaires sociaux.

Pour bon nombre de jeunes, la réussite tant vantée dans une société qui prône l'ascension sociale était un parcours du combattant. Désormais, elle est reléguée à l'espoir incertain. Notre politique publique doit donc être ambitieuse. Mieux, elle doit être la plus optimiste possible, notamment en ce qui concerne la filière d'excellence qu'est l'apprentissage professionnel. Avant la crise sanitaire, les indicateurs étaient au vert. en Île-de-France, près de 90 000 apprentis et préapprentis étaient inscrits à la rentrée 2018-2019. Sur l'ensemble du territoire national, l'année 2020 devait confirmer cette tendance, même s'il était parfois compliqué, pour les apprentis, Cependant, les professionnels du secteur sont actuellement inquiets pour les contrats en alternance lors de la rentrée prochaine. Les effets risquent de se faire sentir, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. J'avais deux questions à vous poser, monsieur le secrétaire d'État. Vous avez déjà répondu à la première, sur l'apprentissage, ce dont je vous remercie. Parallèlement, ne serait-il pas temps de réinventer les emplois d'avenir basés sur une formation professionnelle aussi bien dans le secteur marchand que dans le secteur non marchand ? C'est une demande formulée par les missions locales. En effet, ce dispositif fonctionnait très bien pour une population dite « précaire », car il apportait une formation professionnelle adaptée aux besoins de l'entreprise. La suppression brutale de cette mesure a créé un déséquilibre.

outre ce qui sera annoncé demain sur le soutien aux entreprises et aux centres de formation pour continuer à développer l'apprentissage, nous devons aussi aller chercher les jeunes qui étaient en apprentissage au moment du confinement et qui, pour certains, ont décroché.

de 41,5 % au cours des trois derniers mois. Ce sont évidemment les jeunes de moins de 25 ans qui paient le plus lourd tribut, avec une hausse de 39,5 % de demandes rien qu'en avril. À la même période, en 2019, la mission locale Nice-Côte d'Azur recensait 834 recrutements, alors que 112 seulement seront finalisés cette année, soit une baisse d'insertion professionnelle de 84 % en un an. Du côté de l'apprentissage, la situation n'est pas meilleure : les élèves sont moins nombreux à pouvoir suivre les cours dans les CFA, puisque ces établissements rouvrent à la carte. Autre problème pour les apprentis, cela a été indiqué : leur diplôme est menacé, puisque leur formation pratique a été stoppée ou annulée. De nombreuses entreprises qui les accueillent en temps normal ont été fermées et rouvrent sous conditions. Ces conséquences inquiétantes sur les contrats d'apprentissage se remarquent plus particulièrement dans certains secteurs importants dans les Alpes-Maritimes. Je pense à l'hôtellerie et à la restauration, puisque les offres sont moins nombreuses, alors que 80 % des contrats d'apprentissage courent entre avril et octobre. Monsieur le secrétaire d'État, entendez-vous élargir le fonds d'aide aux jeunes afin de pouvoir apporter un soutien plus durable que l'aide exceptionnelle de 200 euros par jeune qui a été annoncée en mai ? Comptez-vous renforcer les contrats aidés dans le secteur non marchand, notamment au sein des collectivités territoriales ? Enfin, l'emploi des jeunes passera forcément par une baisse des charges. Il faut qu'il y ait une incitation financière. À cet égard, seriez-vous favorable à une exonération des charges pour les entreprises qui recruteraient un jeune en CDI ?

maintenant dans une période trouble sur le marché de l'emploi et pour l'insertion des jeunes. Il faudra un accompagnement plus durable dans ce contexte. Par conséquent, oui, il faut un accompagnement financier renforcé

par toujours plus d'éducation, mais aussi, j'en suis convaincue, par la rencontre avec d'autres cultures, la découverte de l'autre. Malheureusement, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 ont eu un impact désastreux sur la mobilité internationale des étudiants. Si la majorité de ceux qui étaient en échange à l'étranger cette année a pu rentrer avant la fermeture des frontières, l'incertitude est grande pour ceux qui avaient prévu un échange pour la prochaine rentrée universitaire.

nombreuses universités proposeront également des cours en ligne. Les Erasmus+ pourront participer à des mobilités hybrides associant des activités virtuelles avec une mobilité physique à l'étranger dès lors que la situation le permettra. Hélas, il est à craindre que ces cours en ligne ne remplacent jamais les apports résultant de l'immersion dans un autre pays et de la rencontre d'une autre culture. Par ailleurs, de nombreux jeunes qui avaient obtenu un service civique à l'étranger ou un programme vacances-travail ont vu leur projet d'expatriation s'écrouler subitement et se retrouvent bien souvent sans perspective d'emploi. Or ces programmes sont plébiscités par des jeunes qui éprouvent des difficultés à s'insérer professionnellement en France. Monsieur le secrétaire d'État, alors que le risque est grand que l'épidémie de Covid-19 entraîne, un peu partout dans le monde, un repli sur soi, comment comptez-vous donner un nouvel élan à la mobilité des jeunes, bien souvent indispensable pour s'insérer dans la vie professionnelle ?

s'il est un point sur lequel nous nous accordons à 100 %, voire à 200 %, c'est bien celui de la mobilité européenne et internationale des jeunes, qui est à la fois, vous l'avez dit, essentielle pour leur formation, les compétences qu'ils développent et leur insertion dans l'emploi, mais aussi pour la destinée de nos nations et l'avenir de l'Europe. Le Président de la République a fixé un objectif extrêmement ambitieux dans le discours de la Sorbonne : la moitié d'une classe d'âge devra avoir passé au moins six mois dans un autre pays européen à l'horizon de 2024. Il est clair que la situation que nous vivons rend difficile cette mobilisation, mais nous allons poursuivre nos efforts, parce que nous y croyons. J'ai participé voilà deux semaines à une réunion dématérialisée des ministres européens de la jeunesse. Nous nous sommes tous accordés sur cette grande priorité. il faudra immédiatement faire repartir le plus fortement possible le programme Erasmus+, le corps européen de solidarité et tous les dispositifs de mobilité en direction des jeunes. C'est un engagement que je prends ici devant vous. Cela fait partie de nos très grandes priorités. Je disais que les perspectives en

d'une palette que nous allons développer très activement, sur laquelle nous allons investir, une fois que les frontières seront rouvertes, pour permettre à des jeunes d'acquérir des compétences et des expériences qui leur seront utiles lors de leur insertion sur le marché de l'emploi, lorsque les turbulences se seront éloignées.

remercie nos collègues du groupe socialiste et républicain d'avoir organisé ce débat sur les politiques à destination de la jeunesse à mettre en oeuvre au regard de la crise sanitaire qui nous touche et de la crise économique et sociale qui s'annonce. Chaque année, de nombreux jeunes, étudiants ou non, exercent une activité rémunérée leur permettant de vivre de manière autonome. Si le Gouvernement a annoncé une aide de 200 euros aux étudiants précaires et aux jeunes de moins de 25 ans bénéficiant de l'aide personnalisée au logement (APL), force est de constater qu'une partie du public cible ne pourra pas bénéficier de cette aide. Certains jeunes précaires ne sont pas étudiants, certains étudiants précaires ne touchent pas d'APL, étant logés de manière temporaire chez des amis, de la famille ou des connaissances. Il y a des trous dans la raquette. Avec la crise économique et sociale annoncée, il sera de plus en plus difficile, pour ces jeunes précaires, d'accéder à un travail, temporaire ou non, à temps partiel comme à temps complet. Nos jeunes, dans tous les territoires, vont être frappés de plein fouet par cette crise. Il est nécessaire d'anticiper l'avenir. Dans un rapport remis au Premier ministre en mars 2017, Mme Célia Verot et M. Antoine Dulin proposaient la mise en place d'un revenu minimum garanti aux jeunes à partir de leur majorité, ouvert sous conditions de ressources. Ce « revenu socle », limité dans le temps, aurait pour principal atout de ne bénéficier qu'à ceux qui en ont besoin, atténuant les effets de seuil, et de permettre aux jeunes âgés de 18 à 30 ans de bénéficier d'un suivi intensif des services sociaux, veillant à la réussite de leur parcours d'acquisition de l'autonomie et à leur intégration sociale et professionnelle. Monsieur le secrétaire d'État, au regard de la crise qui s'annonce, le Gouvernement compte-t-il travailler sur ce genre de dispositifs d'accompagnement ? Quelles mesures sont envisagées pour permettre aux jeunes les plus précaires, les plus isolés, de ne plus se retrouver en dehors des dispositifs d'aide et, grâce à la solidarité

le 15 avril dernier, Jean-Michel Blanquer, en annonçant le lancement de cette opération, a évoqué à la fois les colonies de vacances, des accueils de loisirs et des soutiens scolaires gratuits pour les décrocheurs. Vous avez vous-même indiqué à l'instant, monsieur le secrétaire d'État, que certains lycées professionnels pourraient rester ouverts. ouverts. Si nous saluons cette proposition, dont l'objectif est de permettre aux élèves de rattraper les lacunes liées à l'enseignement à distance pendant le confinement, nous souhaiterions en connaître les détails. Le confinement a renforcé, je le crains, les inégalités sociales. Tous les enfants n'ont pas vécu de façon identique l'école à la maison. Dans le Nord, par exemple, seulement 20 % des collégiens vont retrouver le chemin de leur établissement scolaire. Les élèves les plus en difficulté ont souvent été injoignables durant cette période et les disparités entre les enfants ont pu s'accentuer. Les collectivités et les professionnels du secteur se tiennent prêts. Ils sont dans l'attente de directives gouvernementales. Il est urgent de définir le rôle des intervenants dans ces colonies de vacances éducatives et leur fonctionnement. Il faudra capitaliser sur nos acquis

pour les jeunes. Ayant vécu une période très difficile de confinement, les jeunes auront peut-être plus que jamais le besoin de s'aérer, de s'évader, d'aller dans la nature, de sortir de chez eux et de leur quartier, d'aller au contact d'autres enfants.

formation. Sans sous-estimer les difficultés que vont rencontrer les jeunes non qualifiés, éloignés de l'emploi et de toute formation, je souhaiterais appeler votre attention sur un public qui n'est traditionnellement pas visé par les politiques publiques de soutien à l'embauche, à savoir les jeunes diplômés à bac+4 et à bac+5 qui vont arriver sur un marché du travail très fortement dégradé. Ces jeunes, qui terminent généralement leur cursus par un stage donnant bien souvent lieu à une embauche, ont été privés de cette chance durant le confinement. À cela s'ajoute bien évidemment la récession importante dans laquelle est entré notre pays. L'absence de visibilité quant à l'avenir a contraint les entreprises à diminuer, sinon à geler complètement leurs embauches. Pour ces jeunes diplômés, le risque de déclassement est important : ne pouvant rester durablement sans revenus, ils pourraient être contraints de se tourner vers des emplois qui ne correspondent pas à leurs compétences ni à leurs qualifications.

du moins pour le service civique. Nous avançons sur deux volets : susciter des offres d'emploi en soutenant les entreprises et permettre aux jeunes d'accéder à des dispositifs utiles pour eux dans l'attente que le marché de l'emploi sorte des turbulences dans lesquelles il est entré.

avant la pandémie de Covid-19, les jeunes étaient déjà les premières victimes de la pauvreté : un jeune sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Demain, ils subiront de plein fouet la crise économique et sociale qui s'annonce, en particulier la hausse sans précédent du chômage.

Pour faire en sorte que certains ne se retrouvent en situation de grande précarité, sans aucune source de revenus, il faut ouvrir le RSA aux jeunes dès 18 ans. Dans les faits, il s'agirait d'un minimum social, un filet de sécurité en somme, qui ne serait accessible qu'à ceux qui sont sans ressources. Dans le même temps, il serait bien évidemment nécessaire de mener des actions ciblées en matière d'emploi, d'insertion, de lutte contre le décrochage scolaire. Muscler, comme vous l'avez déclaré récemment, le service civique ou la garantie jeunes ne permettra pas de faire face aux enjeux humains et sociaux, conjoncturels, résultant de la crise. Monsieur le secrétaire d'État, les grandes associations et collectifs de lutte contre la pauvreté qui oeuvrent en direction de la jeunesse vous alertent. Il y a urgence Dans une société développée prônant l'égalité des droits, il convient de s'assurer de l'égal accès des jeunes à un niveau de ressources minimum. Il ne s'agit nullement, comme vous l'avez dit, de se placer dans un « esprit de défaite », mais bien d'apporter une aide vitale dans un moment de l'histoire exceptionnel à raison de sa gravité. Cet hiver, vous aviez admis que le projet de revenu universel d'activité devrait nécessairement être ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans. Continuez donc sur la voie du pragmatisme et tenez compte de la situation exceptionnelle.

année. Je crois beaucoup à ce dispositif et au Pacea pour accompagner les jeunes financièrement. Ce dispositif représente une aide qui correspond peu ou prou au RSA, mais avec un accompagnement

même si je ne mésestime pas les dispositifs déjà mis en place. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! Il faut une réponse urgente, une réponse concrète, pour ces milliers de jeunes qui se retrouvent sans ressources, sans emploi et en très grande difficulté.

L'apprentissage est l'une des meilleures méthodes pédagogiques pour transférer connaissances et savoir-faire et sans doute aussi le meilleur levier d'insertion des jeunes- 75 %. Les jeunes ont envie de travailler, ils veulent apprendre un métier. Avant la crise sanitaire, la dynamique était réelle. Il faut bien reconnaître que la situation était inédite. Les jeunes sont les premiers touchés par le ralentissement de l'économie. Ils sont inquiets. Les entreprises vont-elles continuer à accueillir des apprentis à la rentrée ? Selon le Medef, il pourrait y avoir « 300 000 potentiels apprentis sur le carreau » en septembre. Les centres de formation des apprentis sont également préoccupés dans la mesure où leur financement dépend du nombre de contrats signés. Monsieur le secrétaire d'État, la crise sanitaire a fait éclater au grand jour la désindustrialisation de la France, ce qui pose des problématiques de pénurie, d'expertise et de qualification. Aujourd'hui, il est essentiel de déployer des solutions en matière de transfert de compétences, de formation et d'attractivité des métiers. Il faut donc investir massivement dans la jeunesse afin de répondre à ses craintes quant à l'avenir. La filière de l'apprentissage attend des mesures fortes du Gouvernement. Quel est votre plan pour relancer l'apprentissage et comment encourager les entreprises à embaucher des apprentis ?

trouvent dans cette voie une manière de construire leur avenir, de se construire et de prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Nous serons au rendez-vous de cette exigence. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour la réplique.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, puisque nous débattons des nouvelles politiques publiques qu'il conviendrait de mettre en place pour aider les jeunes face à cette crise sans précédent, je voudrais aborder la question de la fracture numérique. On croit à tort que l'illectronisme et l'exclusion numérique ne frappent que nos aînés. Grossière erreur Certes, un jeune entre 18 et 24 ans maîtrisera peut-être l'usage des réseaux sociaux sur son téléphone portable, mais cela n'implique pas pour autant qu'il sache naviguer correctement sur un site de l'administration publique ou une plateforme de réservation ni qu'il sache effectuer une recherche efficace sur internet pour s'informer sans être victime de. La crise

Pour les étudiants, le confinement a entraîné une rupture : les cours ont dû être suivis à distance, les ressources en ligne privilégiées et l'aide des professeurs a pu, le cas échéant, s'avérer plus difficile à obtenir. Ce sont les élèves issus de milieux défavorisés qui ont fait les frais de cette distanciation pédagogique. confortables, d'une connexion internet parfois défaillante, ils connaissent les plus grandes difficultés pour étudier ou préparer leurs concours. D'après une étude sur l'école à la maison durant le confinement, 24,3 % des parents d'origine modeste jugeaient leur équipement et leur accès internet insuffisants contre 17 % des familles plus aisées. Les chiffres sont encore plus marquants en ce qui concerne le sentiment de compétence informatique : 45 % des parents des classes supérieures se sentent tout à fait capables de répondre aux exigences techniques numériques de l'école à la maison contre seulement 31 % des parents Face à la nécessité d'avoir au quotidien accès aux outils numériques, que ce soit dans sa vie professionnelle, privée ou citoyenne, cette inégalité numérique est un symptôme de toutes les autres inégalités sociales que connaissent certains de nos concitoyens, voire un facteur aggravant particulièrement inquiétant chez les jeunes. Sachant que près de 20 derniers, par manque de maîtrise, renoncent à faire une démarche administrative sur internet, à envoyer un mail important ou à faire un achat, on comprend que l'illectronisme n'est pas qu'une question de manque d'équipement performant. On observe de la même manière de nombreuses inégalités Réduire cette fracture est un objectif essentiel des politiques publiques, car les inégalités numériques en engendrent d'autres. Il ne sert à rien de distribuer des tablettes aux étudiants si l'on n'intègre pas la formation à ces outils dans la scolarité obligatoire. Monsieur le secrétaire d'État, quelle est votre réponse face à ce défi de société ?

quand on décide de confiner le pays, de fermer les établissements scolaires et que les enfants ne sont plus face aux enseignants, la grande priorité doit être de permettre

généralisé. Nous avons pu proposer cette solution parce que nous avions travaillé avec le CNED depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, pour être capables de réagir immédiatement au cas où surviendrait ce type d'événement. La plupart des autres pays européens

Entre 2018 et 2019, le nombre de contrats d'apprentissage signés a ainsi progressé de 16 %, portant à plus de 480 000 le nombre d'apprentis. Cet engouement s'explique notamment par un taux d'insertion sur le marché de l'emploi des apprentis de près de 75 %, ce qui en fait un puissant levier pour à l'emploi. La crise sanitaire que traverse notre pays est venue compromettre cette amélioration et fragiliser cette voie d'accès particulièrement importante pour l'emploi des jeunes. jeunes. Avec l'arrêt brutal de notre économie, de nombreuses entreprises sont contraintes de revoir- et on peut les comprendre -leurs priorités en matière d'embauche. C'est notamment le cas des PME, des TPE et des artisans, principaux viviers de l'apprentissage.

Malgré le contexte de crise sanitaire, les missions locales sont pleinement engagées dans leur mission à destination des jeunes et je souhaite rappeler qu'elles sont des actrices importantes au plus près du terrain.

À ce jour, elles ont manqué de soutien de leur ministère de tutelle dans le cadre de leur adaptation à l'épidémie de Covid-19 : leurs frais liés à la crise n'ont pas été pris en charge, au seul motif que les missions locales ne sont que délégataires d'une mission de service public. Je souhaitais rappeler cette injustice, monsieur le secrétaire En parallèle, un premier bilan a été établi confirmant le maintien du lien avec les jeunes en cette période. En revanche, on constate une baisse significative, de plus de 50 %, des propositions faites aux jeunes en raison de la fermeture des organismes de formation, des CFA et de la diminution des offres d'emploi. Cette situation doit nous alerter sur les résultats : les indicateurs négociés dans le cadre de la convention pluriannuelle d'objectifs sont, à ce jour, totalement inappropriés. Or le financement est lié à ces mêmes indicateurs de performance qui ne seront évidemment pas atteints en raison de la crise sanitaire.

deux temps et, dans le cadre de la mission d'intérêt général, les jeunes doivent aller dans une association ou auprès d'un corps en uniforme pour apporter leur aide. Nous développerons de grandes causes, en lien avec la crise que nous vivons. Bien évidemment, l'intergénérationnel et le lien avec nos aînés, ainsi que le soutien aux plus vulnérables

plus d'un titre. Tout d'abord, à titre individuel, ils sont le réceptacle indirect et presque mécanique des dommages causés par la crise, singulièrement sur leurs parents.

la demande du groupe socialiste et républicain, d'une proposition de résolution demandant au Gouvernement de mettre en oeuvre une imposition de solidarité sur le capital afin de renforcer la justice fiscale et sociale et de répondre au défi de financement de la crise sanitaire, économique et sociale du Covid-19 présentée, en application de l'article 34-1 de la Constitution, par MM. Patrick Kanner, Vincent Éblé, Claude Raynal, Jacques Bigot et plusieurs de leurs collègues

Madame la secrétaire d'État, votre gouvernement a fait du ruissellement son credo, l'alpha et l'oméga de votre politique non seulement économique, mais aussi sociale. L'idée que, lorsque les pouvoirs publics favorisent l'enrichissement des plus aisés de nos compatriotes, il en découle un effet économique positif indirect pour l'ensemble de la population est une mystification, car personne, jamais, ne l'a observé. Schématiquement, il s'agit de la croyance magique selon laquelle, lorsque l'une des toutes premières fortunes de France gagne 70 millions d'euros, chaque Français en gagne un. Je voudrais tout d'abord m'attarder sur le fondement philosophique de cette théorie. Quand bien même ces résultats seraient assurés, ce qui bien sûr n'est pas le cas, vous ne semblez pas voir, plus précisément vous ne voulez pas voir, l'aggravation des inégalités qui découle inéluctablement d'une telle politique économique.

Il indique que le savoir est objectivement et subjectivement suffisant, quand l'opinion est pour sa part objectivement insuffisante et subjectivement suffisante. Quant à la croyance, elle est objectivement et subjectivement insuffisante.

une certitude économique indépassable. Ce travail a en effet démontré qu'il n'y a pas de ruissellement. Il permet également de mettre en relief une forme d'hypocrisie du Gouvernement en la matière, puisque cet état de fait était déjà révélé à Bercy par le logiciel Mésange et nous avait été communiqué. Ce logiciel ne prévoyait que des résultats très modestes, pour ne pas dire quasi nuls, à long terme, sur vingt ans : hausse de 0,5 point de PIB et création de 50 000 emplois seulement. Ainsi, la théorie du ruissellement n'est plus, madame la secrétaire d'État, qu'une croyance parfaitement insuffisante pour légitimer la conduite d'une politique publique d'allégement constant et déterminé de la fiscalité des Français les plus riches. la réforme fiscale de la loi de finances pour 2018, vous avez prétendu soutenir notre économie nationale. Mais vous avez sorti du champ de l'impôt sur la fortune de nombreux capitaux et actifs, y compris des biens de consommation de luxe tels que yachts, voitures de course, chevaux, métaux précieux, titres de dette souveraine d'États étrangers, soit des objets et matières purement spéculatifs et parfaitement improductifs pour notre économie nationale, alors que, paradoxalement, d'autres capitaux et biens, productifs et concrètement utiles à l'économie et à l'emploi, sont taxés au titre de l'imposition foncière que vous avez créée : il s'agit des locaux industriels et commerciaux, des immeubles de bureaux ou d'habitation. En définitive, l'imposition du capital en France est donc aujourd'hui fondée sur une théorie parfaitement fumeuse et se traduit par un dispositif totalement contradictoire avec l'intention exposée initialement de favoriser notre économie. Aujourd'hui, le Gouvernement nous ayant refusé le bénéfice de l'urgence qu'il s'accorde à lui-même en permanence, finalement une proposition de résolution plutôt qu'une proposition de loi qui nous permet d'échanger sur les principes et les intentions plutôt que sur un dispositif législatif déjà opérationnel. C'est un bien pour un mal, car nous voulons échanger et convaincre à la fois le Gouvernement et la majorité sénatoriale de la nécessité d'une telle réforme. Nous ne souhaitons pas la reproduction de modalités fiscales anciennes. Nous sommes en effet tout à fait disposés à amender et infléchir une nouvelle loi pour un dispositif entièrement nouveau. L'important est de bien considérer les objectifs fixés, car l'acceptabilité est centrale en matière fiscale. C'est d'ailleurs dans cette perspective, et parce qu'il ne doit y avoir ni totem ni tabou en la matière, que nous avons volontairement écarté, mes chers collègues, l'appellation d'impôt de solidarité sur la fortune, qui chagrine certains d'entre vous et présente le risque de laisser croire à un retour en arrière sans rapport avec notre intention.

découlant principalement d'une forte hausse des inégalités patrimoniales. Pas étonnant que, fort de ces analyses, cet économiste fasse partie, avec Esther Duflo, prix Nobel française des personnalités qui appellent de leurs voeux la création d'un impôt sur le capital. J'entends même des voix s'exprimer sur ce thème au sein de votre majorité présidentielle ! Les idées justes ne peuvent pas être écartées d'un revers de la main ou par une simple affirmation idéologique contredite Aujourd'hui mes chers collègues, je vous le dis tel que je le pense, exclure de nos travaux ces questions serait irresponsable. C'est pourquoi, vous le savez, le groupe socialiste et républicain a travaillé ces derniers mois sur des sujets connexes tels que les droits de succession, un ISF 2.0 ou encore les encours d'assurance vie qui découlent ou témoignent, en fonction des points de vue, de la hausse des inégalités. Se pose ainsi la question de rétablir l'équité contributive à l'impôt, gravement mise à mal. Cette nécessité est fortement ressentie, à raison, par nos concitoyens.

est aussi celui des symboles et des mobilisations construites autour des représentations et des convictions. Il est difficile- c'est un euphémisme -de contredire ce ressenti quand on constate les exonérations massives dont bénéficie aujourd'hui le premier décile- et le premier centile -des contribuables français. Le groupe Le groupe socialiste et républicain estime en ce sens que nous avons collectivement, mes chers collègues, le devoir de rétablir une imposition juste et équitable en fonction des ressources réelles de nos compatriotes. Les plus fortunés doivent prendre toute leur part, ni plus ni moins. Cela est particulièrement vrai pour les très, très, très riches, dont la capacité contributive est certaine, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Repenser une imposition de solidarité sur le capital n'est pas une question dogmatique, mais seulement une question de nécessité pour que la solidarité de notre société soit entière, au travers de dispositifs fiscaux plus justes. Ceux qui disent que le produit sera trop faible au regard des besoins du moment se coupent d'une recette utile, car ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et nous dire que « le besoin est de plusieurs dizaines de milliards d'euros, donc une petite recette est insuffisante », c'est de l'idéologie pure Sous prétexte que la recette ne serait comprise qu'entre 3,5 milliards et 5 milliards d'euros, on devrait l'exclure ? Je ne comprends pas cet argument, mes chers collègues. Je le comprends d'autant moins que, à la suite du « grand confinement qu'a connu notre planète, les pouvoirs publics ont un besoin sans précédent de ressources. Or, dans les circonstances actuelles, seul le capital est mobilisable : ni les revenus ni la consommation ne le sont. Rejeter une réflexion sur l'imposition du capital, le stock plutôt que le flux, est un non-sens économique absolu. Ceux-là négligent au surplus la question pourtant essentielle en matière d'équité contributive des représentations symboliques, desquelles découle l'acceptabilité des dispositifs fiscaux. dirai quelques mots sur ce que l'on pourrait imaginer. La nouvelle imposition que nous appelons de nos voeux se fonde sur plusieurs principes. En premier lieu, la progressivité est réaffirmée. Elle permettra de mobiliser le premier centile de manière équilibrée et équitable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cela passerait par la suppression du « plafonnement du plafonnement », comme cela fut proposé par le gouvernement Juppé et validé juridiquement par le Conseil constitutionnel, mais aussi par la définition de barèmes distinguant les « petits » riches, et notamment les personnes pouvant se retrouver dans la situation de la veuve de l'île de Ré, pour reprendre un exemple connu de tous. En second lieu, et je sais toute la vigilance de notre rapporteur général sur ce point, il faut intégrer une distinction entre le capital productif et le capital improductif. Je le dis tel que je le pense : Albéric de Montgolfier a raison sur ce point.

Ce concept nous semble transposable à l'imposition du capital, tout comme les enjeux de la transition écologique. Nous pouvons et nous devons les intégrer à la définition d'une nouvelle imposition sur le capital. La question des nouvelles recettes à trouver ne doit pas nous affranchir d'une remise à plat significative de notre fiscalité, qui craque déjà depuis beaucoup trop longtemps. Au contraire, la situation exceptionnelle que nous traversons nous oblige à être très ambitieux et à aller au bout d'une refonte totale. C'est notre responsabilité, pour ne pas aggraver une situation déjà tendue et éviter de la léguer aux prochaines générations. Le groupe socialiste et républicain souhaite conduire cette réflexion majeure. Tel est l'objet de la proposition de résolution que nous vous soumettons. La

En effet, dans l'euphorie des premiers temps du quinquennat, ce gouvernement avait supprimé l'ISF, pensant ainsi, par cette « courageuse » décision, tirer un trait définitif sur l'idée « saugrenue » de taxer les plus fortunés de nos concitoyens. L'ISF était accusé de faire fuir les riches, privant ainsi nos entreprises de leurs capitaux. Pourtant, aucune étude n'a étayé cette thèse. Entre 2011 et 2017, le nombre de redevables de l'ISF était même passé de 287 000 à 358 000 ménages. Les riches n'ont pas pu revenir, puisqu'ils n'étaient pas partis ! En revanche, alors que l'ISF rapportait 5 milliards d'euros par an à l'État, l'impôt sur la fortune immobilière en a fourni 1,3 milliard en 2019. Comme le Gouvernement a aussi diminué la fiscalité sur les revenus du capital, ce sont 4,5 milliards d'euros qui manquent chaque année dans les caisses de l'État, soit plus de la moitié du budget annuel du ministère de la justice. Durant le confinement, des millions de personnes auront vu leurs revenus s'effondrer. De nombreuses petites entreprises seront malheureusement confrontées à la faillite, leurs salariés se retrouveront au chômage, leurs ex-dirigeants sans revenus. Dans ces conditions, les plus fortunés d'entre nous, rebaptisés à une époque « premiers de cordée », doivent comprendre qu'il est dans leur intérêt de contribuer beaucoup plus fortement et durablement au financement des services publics et de la solidarité, dont ils bénéficient aussi, comme tout un chacun. La crise sanitaire a ébranlé le monde et replacé au coeur du débat politique les questions fiscales, et notamment la fiscalité des gros patrimoines et du capital. Nous le constatons quotidiennement, mes chers collègues, le sujet s'impose. De nombreuses voix s'expriment, provenant d'horizons et de sensibilités très divers : syndicalistes, économistes, philosophes, intellectuels, et également, Vincent Éblé le rappelait, responsables politiques de la majorité présidentielle. Ainsi, M. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, déclarait il y a quelques jours : « S'interroger sur une contribution des plus aisés, pourquoi pas ? les plus riches devraient contribuer davantage », et le président du groupe Modem, soutien de la majorité, M. Patrick Mignola, qu'« il faut créer un impôt sur la fortune improductive

L'ISF, c'est le combat du XX siècle », ou encore : « Rétablir l'ISF serait de la pure démagogie ». Tout Bercy est mobilisé. Madame la secrétaire d'État, je me permets de vous citer : « Avec le retour à l'ISF, on se trompe de combat. Des formules choc, aux mots bien choisis ; mais, au fond, jamais de démonstration étayée ! Ces propos sont doux aux oreilles de nos collègues de la majorité sénatoriale. M. Retailleau déclarait il y a quelque temps : « Je suis contre le rétablissement de l'ISF. » Cela a, au moins, le mérite d'une très grande clarté et d'une grande cohérence. C'est dans ce contexte que nos collègues du groupe socialiste et républicain avancent l'idée d'une imposition de solidarité sur le capital. Exit l'ISF, voici donc l'ISC. Examinons un instant les termes de cette proposition, dont certains, je veux le dire d'emblée, nous laissent un peu sur notre faim. Il en est ainsi du relèvement du seuil d'assujettissement, que vous voulez porter à 1,8 million d'euros. Chacun ici se souvient que le seuil d'assujettissement à l'ISF était, avant 2007, fixé à 800 000 euros

nous partageons donc vos constats, vos propositions nous paraissent malheureusement manquer d'ambition, vu l'ampleur des difficultés qui sont devant nous, tant sur le plan économique que sur le plan social. Faire contribuer les hauts revenus serait de nature à conforter la notion de consentement à l'impôt, afin que chacun contribue « en raison de ses facultés ». Concrètement, il faut que les informations sur les portefeuilles financiers, par exemple, soient transmises automatiquement par les banques françaises et étrangères à l'administration fiscale. Rétablir cet impôt en le rénovant serait aussi un début de réponse à la très forte demande de justice fiscale, et par là même de justice sociale,

Capus. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le rétablissement de l'ISF fait figure non pas de sparadrap, mais de révolution. Cette idée, comme un astre sur son orbite, ressurgit depuis 2017 à intervalles réguliers dans le ciel de notre hémicycle. Elle prend tantôt la forme d'une proposition de loi, tantôt celle d'un amendement au projet de loi de finances, et, aujourd'hui, celle d'une proposition de résolution. révolution », une seule lettre de différence ; mais la différence tient parfois à une seule lettre. Ainsi, après l'instauration de l'IFI en remplacement de l'ISF, il nous est maintenant proposé de passer à l'ISC. Après tout, si les mots comptent, les lettres aussi ! Hier impôt de solidarité sur la fortune, demain, peut-être, impôt de solidarité sur le capital : fortune ou capital, telle est la question. Mais derrière ces mots ronflants, qui sonnent comme des titres de magazines d'actualités économiques, un concept fait son retour : la justice sociale. Qu'est-ce que la justice sociale ? Vaste sujet On peut commencer par dire ce qu'elle n'est pas. Les auteurs de cette proposition de résolution ont ainsi pris soin de la distinguer de la haine des riches. Dans le climat social qui est le nôtre, c'est une précision heureuse, à tout le moins bienvenue. précision ne vaut pas définition, car ce concept est souvent brandi en étendard, mais rarement défini au niveau des principes. Or c'est là tout l'enjeu. La justice sociale ou fiscale ne saurait simplement signifier toujours plus d'impôt pour les riches, et même, parfois, pour les moins riches, comme s'il s'agissait d'une loi analogue à la Les auteurs de cette proposition de résolution en réfèrent à l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Permettez-moi d'en citer la lettre : son article XIII dispose que Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. C'est donc déjà interpréter ce texte que de considérer que l'égale répartition dont il est question justifie la progressivité, d'y voir la justification d'un nécessaire impôt sur les hauts patrimoines en temps de pandémie mondialisée. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne justifie nullement le rétablissement de l'ISF. Il ne s'agit là que d'une interprétation particulière, qui se fonde sur un diagnostic émis sur la société et renvoie à des choix politiques. de même lorsque, une crise sanitaire frappant le pays, le Gouvernement et le Parlement décident de confiner tout le pays quoi qu'il en coûte et d'utiliser l'argent public pour éviter l'effondrement : il s'agit de choix politiques collectifs. En matière de politique fiscale, les choix politiques consistent pour partie à résoudre des équations. Nous venons, au cours de cette crise, pour faire face à l'urgence, de dégrader durablement les comptes publics. Notre taux d'endettement a bondi de 15 points en trois mois- du jamais vu. Nous avons voté l'urgence ; il faut maintenant éviter la dépendance. À cet égard, je me réjouis de trouver dans cette proposition de résolution quelques points de convergence avec les auteurs : l'idée qu'il n'est pas légitime de faire porter le poids financier de cette crise sur nos enfants et nos petits-enfants, et l'idée qu'une taxation accrue de la consommation ou des revenus serait une erreur. Mais, en fixant le même objectif et en cherchant à éviter les mêmes écueils, je ne parviens pas à la même conclusion.

ailleurs, nous ne rembourserons pas notre dette par des taxes symboliques, qui apaisent peut-être des tensions, mais n'améliorent pas vraiment les comptes. Les mesures qui ont été votées depuis 2017 ont considérablement amélioré l'attractivité de la France. Il y a quelques mois encore, les capitaux s'investissaient massivement dans notre pays, le chômage reculait et la croissance progressait. Et si le coronavirus a changé la donne sur le plan économique, il ne contredit en rien la pertinence des choix qui ont été faits. Vous l'aurez compris, mes chers collègues : mon groupe est hostile à l'augmentation des impôts sur le capital, qu'il s'agisse de l'ISF ou d'un ISC. Pour surmonter la crise dans laquelle nous venons à peine d'entrer, nous aurons besoin d'unité nationale davantage que de division ou de boucs émissaires.

Je vous remercie l'initiative de MM. les présidents Kanner et Éblé et de leurs collègues du groupe socialiste, la présente proposition de résolution invite à la création, temporaire, d'un impôt de solidarité sur le capital afin de renforcer la justice fiscale et la justice sociale et de répondre au défi du financement de la crise sanitaire actuelle. Ce nouvel impôt relèverait le seuil d'assujettissement des contribuables de 1,3 à 1,8 million d'euros, ce qui exclurait 40 % des anciens contribuables de l'ISF pour une perte de recettes d'environ 500 millions d'euros, mais pourrait être compensé par un relèvement de deux points du prélèvement forfaitaire unique. Il est également prévu de revenir au « plafonnement du plafonnement » mis en place jadis par le gouvernement Juppé. Le groupe socialiste présente cette proposition de résolution avec l'objectif louable de « sauver le plus de vies possible et préserver notre tissu économique et social, nos emplois et nos entreprises »,

le Président de la République s'était engagé à vérifier en 2020 l'efficacité de l'actuel impôt sur la fortune immobilière : « S'il n'est pas efficace, nous le corrigerons », avait-il dit. nécessaire, tout de même : ni l'éventuelle création d'un impôt de solidarité sur le capital, dont le rendement est estimé à 2,5 milliards d'euros, ni le rétablissement de l'ISF, qui rapporta 4,2 milliards d'euros ni l'actuel IFI, dont le rendement doit atteindre 1,9 milliard d'euros en 2020, ne sont de taille à soutenir le financement de la crise du Covid-19, au titre duquel nous avons déjà voté 110 milliards d'euros de crédits tout aussi indispensables qu'insuffisants au regard des difficultés qui nous attendent. L'ISC est donc plus idéologique que thérapeutique. Il n'empêche qu'il est utile et légitime de s'interroger sur la pertinence de l'impôt sur la fortune immobilière. Succédant à l'ISF, l'IFI a délibérément exclu de sa base taxable les placements bancaires et liquidités, ses concepteurs prétendant ainsi relancer l'investissement dans les entreprises françaises et favoriser la création d'emplois. La commission des finances du Sénat ayant quelques doutes sur l'atteinte de cet objectif, nous attendons avec impatience l'évaluation de l'IFI promise par Emmanuel Macron. Cela dit, le groupe Union Centriste n'a jamais été favorable à l'imposition des seules fortunes immobilières, car les détenteurs d'un patrimoine immobilier ne sont pas plus rentiers que les détenteurs d'un portefeuille d'obligations. Et les premiers concourent parfois davantage à la vitalité de notre économie que les seconds. Par exemple, l'IFI ne taxe plus les valeurs européennes placées dans un plan d'épargne en actions, mais taxe les sociétés d'investissement immobilier cotées qui construisent les centres commerciaux ou encore les sociétés civiles de placement immobilier qui louent des bureaux et des commerces. pourtant, contribue le plus à l'activité et à la création d'emplois ? Qui est, de fait, un pilier essentiel de la filière du BTP ? De notre point de vue, il y a matière à correction. Second point surprenant d'incohérence : l'IFI ne taxe plus le patrimoine polluant. Avions privés, voitures de luxe et yachts ont disparu de la base taxable, alors que le défi écologique est au coeur des préoccupations du Gouvernement.

la question cruciale du financement de la crise sanitaire, il faut d'abord examiner globalement le système actuel. Certaines mesures fiscales adoptées sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, notamment l'institution de la à 30 sur la partie mobilière des revenus de l'épargne et des plus-values, ou encore la réduction progressive du taux de l'impôt sur les sociétés (IS), sont indéniablement positives, en ce sens qu'elles répondent à des distorsions extrêmement coûteuses pour l'économie française. Pour rappel, pendant le quinquennat de François Hollande, l'ensemble des revenus du capital et des plus-values avaient été intégrés aux revenus imposables soumis à la très forte progressivité du barème de l'impôt sur le revenu (IR). Compte tenu des prélèvements sociaux, le taux d'imposition de ces revenus et plus-values pouvait avoisiner 60 %. Il est toujours tentant, politiquement, de s'attaquer au capital déjà constitué mais face à des épargnants de plus en plus informés, de plus en plus réactifs et de plus en plus mobiles, il est vain de penser que l'on peut prélever sur ce stock sans affecter les niveaux de croissance économique et de recettes fiscales. Surtout, la taxation de l'épargne est susceptible de dissuader la formation du capital. Moins de capital signifie une productivité du travail et des salaires réels plus faibles, ou un chômage plus élevé si les salaires réels sont rigides. Il ne faut par ailleurs pas négliger le fait que l'épargne et l'investissement ont des retombées positives sur l'économie, de sorte que les baisses d'imposition associées ne profitent pas qu'aux seuls contribuables concernés. Pour relancer demain l'économie, plusieurs ajustements fiscaux seraient possibles, permettant, à des niveaux de recettes fiscales inchangés, de limiter les distorsions et les dommages infligés à l'économie. La crise du Covid-19 pourrait être l'occasion de « verdir » le système fiscal français en intégrant dans les prix des biens et des services les coûts des dommages causés à l'environnement,

pourrait être mis à profit pour diminuer symétriquement la taxation du travail, voire celle de l'épargne, afin de stimuler l'offre productive. chers collègues, voilà donc quelques contributions à ce débat qui a le mérite de nous faire réfléchir en amont sur les voies possibles d'un financement des réponses à la crise et nous permet de formaliser quelques idées. Notre groupe votera contre cette proposition de résolution, mais soutient cependant l'idée d'une nécessaire révision rapide de l'impôt sur la fortune immobilière.

de transférer l'épargne immobilière, épargne souvent dormante, et ce à long terme, vers l'investissement dans les entreprises, et de participer à la réindustrialisation de notre économie. À l'heure actuelle, les économistes s'accordent à dire qu'il est encore trop tôt pour réellement quantifier les effets de cette mesure. Mais il est certain que cette réforme ne portera pas les fruits escomptés tant que tous les dispositifs allant en ce sens ne seront pas réintroduits. Vous avez d'un côté créé l'IFI, mais, de l'autre, vous avez dissuadé les contribuables de l'impôt sur le revenu de déduire leurs investissements dans le capital des PME. J'y vois une forte contradiction, que je n'arrive toujours pas à expliquer.

mais qui est globalement mal géré, qui s'occupe de sujets qui ne le regardent pas et qui a besoin de se réformer. Certains contribuables se voient prendre plus de 60 % de leurs gains par l'État et- excusez-les -trouvent cela particulièrement injuste. Cependant, n'allez pas caricaturer mon propos en m'accusant d'être anti-impôt, anti-système social, ou contre la solidarité. Loin de là ! Au contraire, même : je suis heureux que nous ayons, en France, des dispositifs qui permettent que les plus aisés viennent en aide aux plus démunis, une assurance santé universelle, l'éducation gratuite pour tous, une défense, intérieure et extérieure, qui a les moyens de nous protéger. Le problème est que l'aide est devenue, en proportion, trop importante, et le régime confiscatoire trop massif, alors même que les redistributions- nous l'avons vu avec l'hôpital pendant la crise sanitaire que nous venons de traverser -sont mal réparties ou, tout simplement, ne sont pas à la hauteur des réalités. La France est le pays le plus taxé de la zone euro, avec un taux de prélèvements obligatoires de 45 % du PIB, pour une dépense publique représentant C'est de la folie ! Pis, seuls 43 % des Français paient de l'impôt, pour une dépense de l'État toujours plus généreuse, le comble de l'irrespect consistant à dire à ces contribuables, comme le font certains, qu'ils ont de la chance d'en payer Face à ce constat, le groupe socialiste et républicain souhaite mettre en place un nouvel impôt qui pèsera sur ceux qui sont déjà les plus gros contributeurs. C'est totalement faux ! Le seul effet de cet impôt sera de relancer le départ des plus riches, entraînant une baisse des recettes et du nombre des contribuables. Plus les contribuables partiront, plus nous serons obligés d'augmenter les taux d'imposition. C'est suicidaire ! Nous sommes au bout d'un système qui est aujourd'hui obsolète. En 2017, quelque 3 800 foyers dont les revenus excèdent 100 000 euros ont quitté notre pays pour partir s'installer à l'étranger. Devons-nous continuer dans cette voie ? Je ne le pense pas. Pouvons-nous nous payer le luxe de laisser partir ceux qui contribuent massivement à la vitalité de notre économie et de nos entreprises ? Je ne le pense pas non plus. Rembourser la dette, objectif vital pour notre économie et pour les générations qui nous succéderont, ne se fera pas par un énième impôt. Il s'agit, aujourd'hui, de créer des richesses et de diminuer nos dépenses, pas de prélever davantage. À rebours des effets que pourrait avoir la mise en place d'un dispositif tel que celui que souhaitent nos collègues socialistes, il serait plus judicieux de s'attaquer enfin au chantier de la reconstruction de notre industrie,

Moins d'impôts, c'est enclencher un cercle vertueux pour notre économie ; plus d'impôts, c'est l'étouffer. Mais accroître les recettes ne sera pas suffisant- je vous l'accorde. L'argent public, l'argent du contribuable, doit être dépensé avec parcimonie et efficience.

qui contribuerait au paiement des charges sociales- c'est ce qu'a fait l'Allemagne, je tiens à le dire. Une telle mesure permettrait de taxer les produits importés tout en déchargeant les produits intérieurs et redonnerait de la compétitivité à nos produits français à faible marge. marge. Il existe de nombreuses pistes pour diminuer le poids de la dette française sans prélever toujours plus sur les entreprises et les ménages. Je suis défavorable au rétablissement de l'ISF, car nous avons besoin des contribuables qui fournissent de l'emploi et de l'activité. Nous devons les inciter à réorienter leur épargne ou leurs investissements vers la réindustrialisation de la France pour rééquilibrer la balance commerciale.

Nous avons besoin de tous les Français, et de tous les contribuables, pour engager la réindustrialisation et sortir de la dette. Dorénavant, nous devons cesser de nous diviser et sortir de cette mise en opposition perpétuelle des riches et des pauvres, des retraités et des actifs, etc. C'est tous ensemble que nous avancerons. Tous les responsables politiques devraient s'accorder sur le postulat suivant : les contribuables, et les Français en général, ne seront plus la variable d'ajustement des dépenses non maîtrisées de l'État.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la crise que nous traversons est sanitaire, économique et sociale. Le rebond que nous appelons de nos voeux doit être rapide, durable et solidaire. Le groupe socialiste et républicain a souhaité débattre sans délai de cette résolution, car nous savons que les crises sont rarement fécondes d'un monde plus juste et qu'un tel accouchement est souvent difficile. La procrastination, en matière de justice fiscale, est une source majeure de frustration. L'idée n'est pas de se bercer d'illusions en imaginant en vase clos un « monde d'après » paradisiaque, mais bien d'agir ici et maintenant. C'est pour cette raison que nous avons inscrit cette disposition à l'ordre du jour de notre assemblée sous la forme d'une proposition de résolution, parce que- le président Éblé

mais espérons que l'idée d'un impôt de solidarité sur le capital fera son chemin et finira par se matérialiser dans la loi, mettant fin à ce nouveau bouclier fiscal instauré par la majorité LR ...

en écartant les petites fortunes immobilières, qui bien souvent, d'ailleurs, n'en sont pas, en nous assurant de la progressivité de ce nouvel ISC et en modernisant les modalités de déclaration, nous avons fait preuve de progressisme. Nous écouterez-vous ? Malheureusement, les déclarations de la majorité sont souvent contradictoires. On sent les tiraillements ! Pour Gérald Darmanin, il y a deux choses à éviter : l'idéologie fiscale et l'augmentation généralisée des salaires, qui tuerait l'emploi. Quand Gérald Darmanin parle d'idéologie fiscale, il parle bien sûr de son opposition épidermique à la réintroduction d'un ISF, rénové ou non. Sur une échelle qui va du président de l'Assemblée nationale au ministre-conseiller régional-maire de Tourcoing, j'ai hâte de voir ou vous vous situez, madame la secrétaire d'État. Je crains d'avoir déjà la réponse, tant la politique du Gouvernement, sur les questions fiscales, est facilement identifiable depuis 2017 : désengagement de l'État et baisse de l'impôt, quel qu'il soit. De là à parler d'idéologie, il n'y a qu'un pas ... Dans votre « nouveau monde », le recul de l'État est érigé en doctrine au profit d'une cause politique. Nous attendons pourtant que vous puissiez vous réinventer.

La réalité qu'occulte le Gouvernement, c'est que ce niveau de prélèvements est lié à un périmètre d'intervention de l'État plus large que chez nos voisins- c'est vrai. C'est une question de choix de société ! Oui, l'État-providence a un coût,

Elle l'a été durant le confinement, elle l'est durant le déconfinement, elle le sera pour faire face aux conséquences sociales de la crise, qui sont devant nous. Vous le savez : vous ne pouvez plus fonctionner avec le logiciel libéral du début du quinquennat ; si vous persistez, nous courons à la catastrophe. Vous ne pouvez plus alléger la fiscalité des plus riches en prétextant un niveau de prélèvements obligatoires trop élevé et supprimer des politiques à destination des plus modestes pour équilibrer les comptes publics- je pense à la réforme de l'aide personnalisée au logement ou à celle de l'assurance chômage.

tout en améliorant, bien sûr, cet impôt. Avec cet impôt de solidarité sur le capital, nous proposons un dispositif qui n'est pas confiscatoire et qui permet à chacun de contribuer à l'effort national selon ses moyens. Les temps qui s'annoncent sont durs il faut tout faire pour empêcher le creusement des inégalités. Notre contribution est modeste, mais indispensable pour permettre à un grand nombre de Français de ne pas basculer dans la précarité. Si cette main tendue est à nouveau rejetée par l'exécutif, les jours qui nous attendent n'auront rien d'heureux.

avait restreint, mais non supprimé, l'impôt sur la fortune, conformément à l'annonce faite par Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale. En remplaçant l'ISF par un impôt sur la seule fortune immobilière, l'IFI, et en instituant un taux fixe d'imposition des revenus du capital, le prélèvement forfaitaire unique ou, fixé à 30 %, le Gouvernement a remis au goût du jour des questions que nous avions dû traiter lors des débats sur le bouclier fiscal, en 2007, lorsque fut supprimé l'impôt sur les grandes fortunes, à l'époque de la première cohabitation ... L'imposition de la fortune fait partie de ces politiques à forte teneur symbolique qui devraient permettre, à première vue, de distinguer la droite et la gauche, selon une ligne en apparence simple. Bien sûr, les choses sont beaucoup plus complexes en réalité. Les controverses sur le bien-fondé économique ou moral de l'ISF ne datent pas de l'élection d'Emmanuel Macron ; elles ont toujours plus ou moins existé. Vous le savez, le radicalisme dont nous nous réclamons s'articule autour de grands principes qui ont façonné la République, tels que la défense des libertés, l'égalité, l'union nationale, la laïcité, la protection de la propriété individuelle ... C'est pourquoi il se reconnaît moins dans les débats souvent teintés de présupposés idéologiques, comme celui de l'imposition de la fortune. Il défend néanmoins le principe de l'impôt, qui doit être acquitté en fonction des capacités contributives de chacun, en accord avec l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il reste attaché à l'idée citoyenne d'un impôt sur le revenu, chère à Joseph Caillaux, alors que notre système fiscal s'est grandement complexifié depuis son instauration voilà un peu plus d'un siècle. Que dire donc de l'établissement d'une imposition plus forte sur le capital ? L'impôt sur la fortune tel qu'il existait jusqu'en 2017 rapportait un peu plus de 4 milliards d'euros par an. On pourra juger que ce n'est pas un montant seulement symbolique, bien qu'il ne représente qu'une petite fraction des recettes publiques. Sa transformation en impôt sur la seule fortune immobilière a surtout révélé la part prépondérante du patrimoine financier chez les ménages les plus aisés. C'était d'ailleurs la volonté du Président de la République de soutenir ce type de patrimoine, jugé davantage productif. Depuis, les oppositions de gauche- socialistes, France insoumise, communistes ... -n'ont eu de cesse de demander le rétablissement d'un impôt sur le patrimoine plus ou moins comparable à celui qui existait avant 2018. C'est également une demande importante du mouvement des « gilets jaunes », qui a eu pour origine une révolte contre un sentiment plus général d'injustice fiscale et sociale. Face à ces revendications, le Gouvernement s'est jusqu'à présent toujours refusé à remettre en question cette réforme, parmi les premières mises en oeuvre au début du quinquennat et qui reste un jalon important de sa politique, malgré le besoin de trouver de nouvelles recettes publiques pour couvrir les dépenses très importantes décidées pour faire face aux conséquences économiques des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19. La commission des finances du Sénat a rendu au mois d'octobre 2019 un intéressant rapport d'évaluation de la transformation de l'ISF en IFI et de l'instauration du PFU, qui a conclu à une certaine précipitation de la réforme et à des effets négatifs insuffisamment pris en compte. Au-delà des idéologiques, c'est effectivement la critique qu'on pourrait formuler n'aurait-il pas mieux valu préparer une réforme plus nuancée, moins empressée, de la fiscalité du patrimoine et en permettre une évaluation réellement efficace ? Rappelons qu'une grande partie des Français s'acquittent déjà d'impôts sur la détention de capital : les taxes foncières. Dans cette perspective, l'IFI ne s'apparente qu'à un impôt additionnel à la taxe foncière pour les patrimoines les plus élevés. Cette réforme semble avoir eu un effet positif sur l'attractivité du pays, comme en témoigne le retour d'un certain nombre de contribuables. En outre, la perte de recettes fiscales n'a pas été aussi forte qu'annoncé. Toutefois, peut-on aller jusqu'à attribuer les bons résultats économiques de la France pendant les trois premières années du quinquennat à cette réforme particulière ? Ne faut-il pas y voir aussi l'effet de réformes antérieures ou intervenues dans des domaines plus structurels, comme la réglementation en matière de droit économique et de droit du travail ? Le doute est permis. Depuis Depuis le 17 mars 2020, le contexte a radicalement changé. Il s'agit non plus de favoriser l'attractivité ou d'améliorer la compétitivité de notre économie, mais de soutenir les entreprises face à une crise majeure et de sauver notre tissu économique des conséquences dramatiques des mesures d'urgence mises en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Hier, le ministre de l'action et des comptes publics a annoncé un chiffre actualisé du déficit public, désormais estimé à 220 milliards d'euros pour 2020 ! Cette dégradation sans précédent des comptes publics va entraîner un endettement record et- hélas ! -probablement le besoin de dégager de nouvelles ressources. Se pose alors la question de la contribution des différents secteurs de la société au redressement économique du pays, en particulier le rôle des plus aisés, et sur la manière la plus adéquate de contribuer. Du strict point de vue des finances publiques, l'imposition du capital peut dégager quelques milliards d'euros de recettes. C'est une contribution, certes, limitée face à l'ampleur de la dépense, mais, là aussi, symbolique. Le relèvement du seuil d'assujettissement de 1,3 million d'euros à 1,8 million d'euros, afin de sortir de l'impôt les « petites fortunes » immobilières, comme le proposent nos collègues socialistes, serait une bonne chose. En effet, depuis l'instauration de l'ISF, le patrimoine moyen des Français a très sensiblement augmenté. La modernisation des modalités déclaratives est aussi une exigence, car c'était un des principaux défauts de l'ISF. Elle reste toutefois à préciser. Force est de constater que les mesures d'urgence sanitaire n'ont pas affecté tous les ménages et toutes les professions de la même manière. C'est pourquoi une taxation du capital ne serait pas moins légitime qu'une taxation accrue de la consommation ou des revenus. La situation des finances publiques sera un sujet de préoccupation encore plus majeur dans les prochains mois. C'est pourquoi les propositions dans leur diversité sont bienvenues. Les membres du groupe du RDSE, dans leur majorité, voteront donc en faveur de cette proposition de résolution ; les autres s'abstiendront.

à l'occasion de la crise des « gilets jaunes » à quel point il était compliqué d'utiliser le levier fiscal en faveur de l'écologie tout en ménageant le pouvoir d'achat. Cet enjeu est devant nous. Par conséquent, si nous voulons, dans la perspective d'échéances politiques futures,

Face à la crise sociale qui vient, la France doit apporter une réponse de justice fiscale, afin de corriger les inégalités, qui se sont creusées au cours des dernières décennies et qui ne cessent de s'aggraver. Face à une société fracturée, où les services publics ont déserté les territoires, où les salaires stagnent et où la précarité s'intensifie, nous avons un devoir politique et quasiment moral : réintroduire dans notre système fiscal un impôt de solidarité sur le capital ou la fortune,

S'il vous plaît, participez au fonds de solidarité. S'il vous plaît, investissez dans l'économie productive. Et merci pour Notre-Dame ! » Mais, mes chers collègues, la différence entre l'impôt et la philanthropie, c'est ce petit détail qu'on appelle la démocratie. Ce sont les élus du peuple qui décident

Nous sommes favorables à l'idée de trois économistes français, Gabriel Zucman, Emmanuel Saez et Camille Landais, qui ont proposé la création d'un impôt européen sur le patrimoine. Cet impôt progressif sur la fortune, qui serait limité dans le temps et à l'échelle européenne, s'appliquerait aux patrimoines de plus de 2 millions d'euros. Ben voyons sortir de la logique unique de solidarité entre les États ; insister sur la solidarité entre les Européens ; ouvrir le débat sur l'instauration d'une véritable et efficace instance démocratique pour gérer les transferts financiers entre États.

Il serait peut-être intéressant de voir comment faire. Mme Pénicaud a récemment demandé aux Français de sortir pour consommer cette épargne. Quelle erreur ! Le monde d'après doit être non pas celui de la relance par la société de consommation, qui mène notre planète à sa perte, mais celui de la résilience par le partage des richesses. Il nous faut comprendre la justice fiscale non comme une règle moralisatrice, mais comme un ciment social. L'avenir de notre pays repose sur le triptyque : justice sociale, démocratie renouvelée et écologie. Pour fonctionner, ce triptyque doit être assis sur un système fiscal juste. C'est le sens de cette proposition et des nombreuses autres que nous formulons.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, l'épidémie que nous traversons est d'une extrême gravité. C'est pourquoi nous avons réagi avec un dispositif puissant, afin d'aider les Français et les entreprises à passer le cap.

Pour ce faire, vous proposez au Gouvernement de mettre en oeuvre une imposition de solidarité sur le capital, voire le rétablissement pur et simple d'un succédané d'ISF. S'il y a bien une leçon que nous devons tirer de cette crise, c'est que les anciennes recettes n'ont pas de raison de fonctionner mieux maintenant qu'avant. Vous avez mal écouté ! Et gardons-nous de parler d'économie ultralibérale dans un pays où l'impôt représente près de la moitié de la richesse créée chaque année et où, aujourd'hui, en tout cas au mois d'avril, près d'un salarié sur deux

du capital utilement mis au service des salariés et des investissements ? Dans le cadre du plan de relance, il paraît évident que nous aurons besoin de trouver des outils pour relancer l'investissement. Il serait contradictoire, dans le même temps, de revenir en arrière en matière de réformes visant à rediriger le capital vers les entreprises. Enfin, je veux dire un mot des inégalités. Les études économiques et sociologiques montrent que la France est l'un des pays où les politiques publiques corrigent le plus fortement les inégalités de revenus, en réduisant les écarts par une redistribution importante en direction des plus modestes- je fais référence

Le combat, c'est l'école, la santé, l'emploi dans les quartiers populaires et les zones rurales, autant de sujets que nous avons pris à bras-le-corps avec le dédoublement des classes en REP et REP+, le plan Pauvreté, le plan Ma santé 2022 ou, dans un autre registre, les territoires d'industrie ou le plan Action coeur de ville. Nous pouvons certainement

J'ajoute que nombre de pays ont de meilleurs résultats en matière d'inégalités avec un niveau de prélèvements bien moindre. Cela relève du savoir et non de l'opinion, pour reprendre vos mots, sénateur. J'aimerais revenir sur la réforme de la fiscalité du capital menée par le Gouvernement. Clairement annoncée par le Président de la République, son objectif était d'améliorer la lisibilité, la prévisibilité et la compétitivité de notre fiscalité,

que chez nos partenaires européens. Chacun peut comprendre que, pour des populations très mobiles, et un capital qui l'est tout autant, cette situation nuisait à l'attractivité de notre pays, donc à l'activité économique et, par suite, à notre situation sociale, à notre préférence pour le chômage et à l'état de nos finances publiques. Ce constat n'a pas changé. Il est même d'autant plus important que nous traversons la plus grave crise économique que connaît notre pays depuis presque un siècle et que nous allons devoir relancer notre économie. La réforme que nous avons réalisée est efficace ; elle a permis à la France de renforcer sa compétitivité et son attractivité. Vous l'avez signalé, les expatriations de contribuables ont ralenti. Les départs de contribuables à l'impôt sur la fortune en 2017 ont été divisés par trois. En 2018 et en 2019, la France a été la première destination européenne en termes d'investissements industriels et de recherche et développement. Notre politique fiscale est clairement ressortie comme un élément expliquant ce regain d'intérêt. Ensuite, cette réforme est équilibrée. Nous n'avons pas touché à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, parce que nous pensons qu'il est légitime que les contribuables les plus aisés contribuent de façon spécifique. L'ISF était un impôt dont le poids baissait relativement quand la richesse augmentait, ce qui est assez paradoxal pour un impôt supposément progressif. L'ISF taxait finalement moins les plus hauts patrimoines que les patrimoines moins élevés, du fait du dispositif de plafonnement de l'ISF en fonction du revenu.

Le Gouvernement a en effet choisi de conserver une réduction d'IFI au titre des dons., les experts du Comité d'évaluation indépendant s'accordent pour dire que le nouveau régime fiscal qui s'applique à l'épargne des ménages avec le PFU et l'IFI est plus simple et plus lisible que le précédent. Ils indiquent également que le nouveau régime dissuade par ailleurs les comportements d'optimisation fiscale, qui étaient en effet induits par le plafonnement, et qui nuisaient non seulement aux recettes publiques, mais aussi à la vie des entreprises, notamment dans les situations de transmission. réforme a vocation à contribuer à réorienter l'épargne des ménages vers l'investissement productif et le financement des entreprises, chose dont nous avons grand besoin aujourd'hui. J'entends vos propositions, madame Vermeillet,

Vous arguez de la nécessité d'une réforme de l'imposition du capital en raison des inégalités et des injustices fiscales subies par les Français, et vous avancez notamment la dimension symbolique de l'ISF. Plutôt que des symboles, je crois que nos concitoyens attendent des faits. Permettez-moi de vous rappeler que les baisses d'impôts engagées sur l'ensemble du quinquennat devraient atteindre 27 milliards d'euros pour les ménages et 13 milliards d'euros pour les entreprises. Concernant l'impôt sur le revenu, nous avons proposé une baisse de 5 milliards d'euros, qui allégera substantiellement l'effort fiscal des classes moyennes et populaires. Ce sont ainsi 17 millions de foyers fiscaux qui connaîtront une diminution de leur impôt sur le revenu, pour un gain moyen d'environ 300 euros. Le gain sera

Nous avons également décidé de reconduire pour 2020 la prime exceptionnelle exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 1 000 euros. Entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, elle a été versée dans près de 400 000 établissements

la redistribution, et ce ne sont là que certains des nombreux dispositifs mis en place pour aider nos concitoyens des classes populaires et moyennes, avant même que la crise ne les frappe. Quant à la CRDS, madame Taillé-Polian, je veux rappeler que c'est l'impôt dont l'assiette est la plus large, puisqu'il s'applique aussi à la vente de bijoux ou de yachts. Utiliser

Pour faire face à la crise, nous avons mené une action puissante et sans équivalent dans notre histoire récente. Rien que pour le plan de soutien, nous avons mobilisé 110 milliards d'euros, dont l'essentiel est est destiné aux salariés grâce au chômage partiel et aux indépendants, commerçants et artisans qui ont été les plus exposés, notamment avec le fonds de solidarité. Dans la balance, vous proposez une réforme symbolique qui permettrait de dégager, selon les calculs, 2,5 milliards d'euros. De notre côté, nous mobilisons 18 milliards d'euros pour le tourisme, 8 milliards d'euros pour l'automobile et les milliers d'emplois qu'elle représente. Nous nous battons aussi pour le secteur aéronautique,

Comment relance-t-on notre économie ? Comment relance-t-on notre industrie ? Comment accélère-t-on les transitions numériques et écologiques ? Comment renforce-t-on notre attractivité et, finalement- le mot est lâché -, notre compétitivité ? Comment

mécanisme d'inclusion carbone aux frontières de l'Union européenne, taxation minimale des entreprises, dans le droit fil des travaux de l'OCDE, ou encore lutte contre la fraude fiscale, notamment en matière de TVA. Ce sont autant de combats que nous avons engagés et que nous poursuivrons activement dans les semaines qui viennent.